La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 18 octobre 2017 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté.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

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les arboriculteurs des Alpes-de-Haute-Provence ont subi, en avril dernier, deux épisodes de gelée noire particulièrement dévastateurs. La capacité de production pour la période 2017-2018 est ainsi gravement affectée. Pour ces agriculteurs, l'enjeu est de préserver une trésorerie suffisante pour pouvoir maintenir leur activité et donner une visibilité aux employés et aux clients, mais aussi aux banques et aux structures de financement de ces exploitations agricoles. Or les procédures d'indemnisation des agriculteurs concernés qui doivent permettre de passer ce cap très difficile ne prennent en compte qu'une petite partie des préjudices subis. En effet, l'arrêté du 17 septembre 2010, qui pose le cadre général des conditions d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents, prévoit des taux d'indemnisation par type et volume de pertes qui ne correspondent pas à la réalité des dommages supportés lors de ces deux épisodes de gelée noire. Je me permets de rappeler, monsieur le ministre, que des dispositions exceptionnelles ont déjà été mobilisées lors d'épisodes similaires pour d'autres départements. L'arrêté du 1 juin 2013 portant modification du taux d'indemnisation applicable aux pertes supérieures à 80 %, à la suite du gel des 16 et 17 mai 2012, a ainsi prévu que, pour une tranche de perte supérieure à 80 %, le taux d'indemnisation de base soit porté à 50 % au lieu de 35 %. Compte tenu de la gravité de ces épisodes et de l'importance de la filière arboricole pour l'ensemble du département des Alpes-de-Haute-Provence, je demande que, de manière similaire, ce taux d'intervention soit augmenté à hauteur de 50 % pour

Ils n'ont pas de répit. Ma question, monsieur le ministre, est la suivante : entendez-vous relever le taux d'indemnisation de ces agriculteurs ; comment comptez-vous accélérer les procédures d'indemnisation ? La parole

Afin d'accompagner les exploitants qui connaissent des difficultés économiques en cette période, plusieurs dispositifs peuvent d'ores et déjà être utilisés : le recours à l'activité partielle pour leurs salariés un dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti pour les parcelles touchées par le gel ; un report du paiement des cotisations sociales auprès des caisses de mutualité sociale agricole. Pour la filière arboricole, les pertes de récolte et de fonds sont éligibles au régime des calamités agricoles. Le travail de reconnaissance au titre des calamités agricoles est en cours au niveau départemental et la majorité des dossiers devrait être examinée au prochain comité En ce qui concerne le taux d'indemnisation en arboriculture, l'arrêté du 17 septembre 2010 prévoit déjà un taux évolutif, compris entre 20 % et 35 %. À ce stade, le Gouvernement n'envisage pas de majorer ce taux. Pour autant, monsieur le sénateur, face à la multiplication

plus largement leurs productions, à travers le dispositif d'assurance récolte contre les risques climatiques. L'État accompagne ces dispositifs assurantiels par une prise en charge partielle des primes ou cotisations d'assurance

pour abaisser la franchise. Des travaux ont été engagés avec les organisations professionnelles agricoles, en particulier les professions viticoles et arboricoles, ainsi qu'avec les assureurs,

En effet, ces produits, qui sont indispensables au traitement des vergers labellisés biologiques, sont homologués par l'Union européenne conformément au cahier des charges qui limite notamment l'emploi des intrants. C'est ainsi que la bouillie sulfocalcique et le Neemazal sont largement utilisés par les arboriculteurs allemands, suisses ou italiens et que nous consommons en France, sous le label bio, des pommes issues de ces vergers. Or, en France, ces agents de base font l'objet d'une dérogation annuelle délivrée par votre administration, sous couvert de la direction générale de l'alimentation. cette dérogation, limitée dans le temps et renouvelable sous certaines conditions, s'appuie entre autres sur le principe de précaution en raison de données toxicologiques. Il n'existe Il n'existe pas de produit de substitution pour lutter efficacement contre les pucerons des arbres fruitiers, si bien que, sans ces produits de base, la pérennité de l'arboriculture bio n'est pas assurée Dans ce contexte, alors que les principes actifs sont connus et que toutes les garanties sont prises, je vous sollicite, monsieur le ministre, pour que de nouvelles dispositions soient mises en oeuvre pour aligner la réglementation française sur celle des autres États membres de l'Union européenne. Je souhaite ainsi que la bouillie sulfocalcique et le Neemazal soient enfin homologués de manière permanente au titre des produits conformes à l'agriculture biologique.

Le Neemazal est un produit phytopharmaceutique à base d'azadirachtine, qui est une substance extraite du margousier. Il s'agit d'une substance active, approuvée en 2011 par l'Union européenne. L'azadirachtine a des propriétés insecticides, qui présentent un intérêt en arboriculture fruitière, en particulier pour lutter contre le puceron cendré, et en culture légumière ou ornementale. Du fait de son origine naturelle, cette substance est utilisable en agriculture biologique. Six demandes d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques à base de cette matière active ont été déposées à l'ANSES. Leur évaluation est en cours et s'approche de son terme. Des décisions relatives à ces demandes d'autorisation de mise sur le marché sont donc attendues en 2018. Afin de répondre à certaines situations d'urgence phytosanitaire dans les vergers de fruits à pépins ou à noyaux et d'agrumes, situations qui ont été signalées depuis 2014, le ministère de l'agriculture a délivré des autorisations dérogatoires d'une durée de 120 jours

bouillie communément appelée bordelaise -, qui présente un caractère de persistance marqué dans l'environnement. La plupart des préparations soufrées sont autorisées en agriculture biologique. À ce jour, une seule firme a montré de l'intérêt pour distribuer en France une préparation Cependant, elle a décidé de soumettre, dans un premier temps, une demande d'autorisation de mise sur le marché en Espagne et de solliciter, ultérieurement, une autorisation en France par la voie de la reconnaissance mutuelle. Selon les dernières informations disponibles, l'examen du dossier en Espagne n'est pas encore

Comme vous le savez, l'arboriculture est déjà durement frappée par des crises structurelles et conjoncturelles et de nombreux professionnels, dont ceux des Hautes-Alpes ou des

très préjudiciable à la production française, à la filière pomme-poire en particulier. La parole

Madame la ministre, le nouveau dispositif de délivrance des cartes d'identité, issu de la réforme Préfectures nouvelle génération, a été généralisé au mois de mars 2017. Actuellement, seules 2 088 communes sont dotées du dispositif de recueil- le DR -et donc habilitées à délivrer les cartes d'identité. Après plusieurs mois de mise en oeuvre et d'observations faites sur le terrain, je pense que cette situation ne peut pas rester figée indéfiniment et qu'il convient d'envisager des évolutions pour tenir compte, d'une part, de la spécificité des territoires et, d'autre part, de l'évolution de l'organisation territoriale.

Une approche objective, prenant en compte les temps de trajet et les difficultés d'accès, justifierait que ces communes soient autorisées à délivrer les cartes d'identité. de l'évolution de l'organisation territoriale, des communes rurales ont fait le choix, parfois difficile, de se regrouper au sein d'une commune nouvelle pour optimiser leurs compétences et mutualiser leurs moyens. évolution territoriale modifie le contexte local et confère désormais à ces communes nouvelles une vocation d'offre de services, qui justifierait qu'elles délivrent les cartes d'identité. dans un contexte où la ruralité a besoin de messages positifs de l'État, j'espère que vous pourrez répondre favorablement à ma demande, qui est simplement fondée sur le bon sens venu du terrain. La parole

Ainsi, les données personnelles sensibles recueillies lors de la constitution des dossiers doivent transiter par des réseaux informatiques dédiés et sécurisés, comme pour les demandes de passeport. Dans un rapport publié en juin 2016, l'Inspection générale de l'administration avait calculé le nombre de dispositifs de recueil supplémentaires qu'il convenait d'installer pour assurer une capacité annuelle de production satisfaisante, dans le respect de l'égalité des territoires.

Les préfets ont été informés, en juillet, de la répartition par département de ces stations biométriques qui a été décidée en considération du taux d'utilisation des stations existantes et de la fréquence des délais de rendez-vous supérieurs à 30 jours. Dans les départements répondant à ces critères, il appartient aux préfets, en concertation avec les associations départementales des maires, de répartir ces nouveaux dispositifs. Dans le Cantal, le taux d'utilisation peu élevé des dispositifs installés ainsi que l'existence de délais de rendez-vous dans les mairies satisfaisants ont amené le ministère à reconduire le dispositif existant.

Cela dit, à l'heure actuelle, comme je vous l'ai indiqué, le système a été reconduit dans le Cantal. Toutefois,

prise des empreintes digitales. En outre, un dispositif de recueil mobile a été mis à la disposition des mairies dans chaque département, afin notamment de recueillir, de manière

sur des territoires à faible démographie, les vastes espaces entraînent des temps de transport très longs et des difficultés d'accès. Je suis de ceux qui pensent que la seule politique efficace et juste d'aménagement du territoire est celle qui prend en compte la diversité et apporte des réponses différenciées.

pour le culte catholique, dans les trois départements d'Alsace-Moselle, les frais de logement du prêtre desservant et de réparation du presbytère sont répartis entre les conseils de fabrique dont le desservant a la charge et donc, indirectement, entre les communes concernées. Dans la même logique, quelles sont les règles applicables pour les frais de logement, de fonctionnement et de réparation du logement d'un rabbin ou d'un pasteur protestant Le cas échéant, je souhaite savoir quels sont les critères administratifs précis de délimitation du ressort territorial à prendre en compte pour définir les communes concernées par la répartition. Par ailleurs, des interrogations du même type se posent au sujet de la répartition des dépenses de grosse réparation des temples protestants et des synagogues. Cette problématique a été évoquée en détail dans la question écrite n° 440 du 13 juillet 2017, posée par mon collègue Jean Louis Masson. Malheureusement, cette question n'a toujours pas obtenu de réponse de votre part. Or il y a un vide juridique, car les fabriques catholiques n'ont pas d'équivalent pour les cultes protestant et israélite. Lorsque des travaux doivent être réalisés dans un temple ou une synagogue, je souhaite savoir si seule la commune d'implantation doit assurer le financement ou si celui-ci incombe à l'ensemble des communes concernées. Le cas échéant, je souhaite connaître le critère administratif précis qui délimite les communes concernées. La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur. Madame la sénatrice, s'agissant des frais de logement des ministres du culte d'Alsace-Moselle, il convient tout d'abord de rappeler que les communes ont la charge exclusive du versement d'une indemnité de logement, en l'absence de presbytère ou de logement mis à disposition par ces communes. Ces modalités sont précisées par l'ordonnance royale du 7 août 1842 relative à l'indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite, qui prévoit l'intervention du préfet de département pour déterminer le montant de l'indemnité due, ainsi que la répartition de cette charge entre les communes bénéficiant de la desserte cultuelle. En revanche, les frais d'entretien de ces bâtiments, lorsqu'ils sont mis à disposition des ministres du culte par les communes, ainsi que des édifices du culte, en général, incombent à titre principal aux établissements publics du culte, à savoir, selon chaque culte, la fabrique d'église, le conseil presbytéral ou le consistoire israélite départemental. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance de ressources de ces établissements publics que les communes composant la circonscription religieuse correspondante sont appelées, à titre subsidiaire, à participer à cette charge, en application de l'article 2543-3 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne le culte catholique, les modalités de cette intervention communale sont précisées par l'article 4 de la loi du 14 février 1810, selon une clé de répartition « au au marc le franc », c'est-à-dire au prorata des contributions directes locales de chacune des communes comprises dans le ressort paroissial. Cependant, aucune disposition équivalente ne s'appliquant aux autres confessions, en particulier au culte protestant pour lequel les communes comprises dans le ressort paroissial n'ont pas été précisément désignées, il est communément admis que pouvait être appliquée, par analogie, la règle de répartition des charges selon le critère fiscal de la loi de La fixation des ressorts rabbiniques a, en revanche, fait l'objet de mesures réglementaires permettant d'identifier le cas échéant les communes appelées à participer à ces frais.

On ne peut donc délibérer sur le choix de la reprise, sans être d'accord au préalable sur l'intérêt communautaire, qui lui-même peut supposer une restitution partielle de la compétence. En outre, un

La parole est à Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur. Madame la sénatrice Loisier, les délais pour harmoniser la compétence scolaire à la suite de la fusion de deux communautés de communes au sein d'une nouvelle intercommunalité sont distincts selon que la compétence est facultative ou optionnelle. Dans le cas de compétences facultatives, comme le sont les services en matière scolaire, une nouvelle communauté de communes dispose d'un délai de deux ans pour conserver ou restituer la compétence. En revanche, pour les compétences optionnelles- dans le domaine scolaire, il s'agit des bâtiments -, ce délai est seulement d'un an. Si elle décide de conserver la compétence optionnelle, la communauté de communes doit ensuite décider de l'intérêt communautaire de la compétence dans les deux ans qui suivent la date de son arrêté de fusion. Jusqu'à la prise de la délibération actant l'intérêt communautaire, et dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la fusion, un exercice territorialisé temporaire de la compétence « bâtiments scolaires » peut être admis. Au-delà de ce délai, la Au-delà de ce délai, la définition de l'intérêt communautaire permet à la nouvelle communauté de communes de déterminer les composantes de cette compétence qui seront exercées à son niveau. jusqu'à la définition de cet intérêt communautaire, et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion, l'intérêt communautaire qui était défini au sein de chacun des anciens établissements

il est conseillé au conseil communautaire de prendre une décision de restitution de compétence avec une date d'entrée en vigueur différée. Cette formule, qui s'applique également en cas de restitution de la compétence en matière de service des écoles, paraît répondre

que les communes décident ultérieurement de transférer de nouveau la compétence à la nouvelle communauté de communes. La parole

notamment quand on doit prendre en compte aussi le calendrier scolaire pour éviter de déménager des enfants et des équipes pédagogiques en cours d'année. La

dans le système d'admission post-bac, dit APB. Ce portail centralisait jusqu'à présent l'ensemble des démarches d'inscription dans l'enseignement Depuis la mise en place du système d'orientation des bacheliers vers différentes formations proposées au niveau supérieur, la complexité et l'opacité du système sont régulièrement critiquées. Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur a présenté au mois de juin dernier un rapport dans lequel il souligne la nécessité d'améliorer l'information des familles sur la procédure et rappelle que « l'algorithme utilisé doit être transparent pour tous

Le Gouvernement a déjà annoncé la fin du tirage au sort pour l'an prochain. La procédure d'admission changera de nom et continuera à utiliser un algorithme.

Je souhaite donc savoir, madame la ministre, quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour rendre la procédure d'admission post-bac transparente et conforme à la loi Informatique et libertés, qui dispose : « Aucune [ ...] décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé

Deseyne, dans une décision rendue publique le 25 septembre dernier, la CNIL a fermement critiqué, devant les difficultés rencontrées pendant la campagne 2017 d'APB, l'absence d'un traitement personnalisé et humain des étudiants, ainsi que le manque d'information des lycéens sur le respect des droits qui leur sont reconnus par la loi Informatique et libertés de 1978. La CNIL confirme donc le constat fait par le Gouvernement dès le mois de juillet dernier le système APB, tel qu'il est conçu actuellement, est un immense gâchis et ne peut plus répondre de manière satisfaisante à l'enjeu que représente l'accès à l'enseignement supérieur pour les futurs étudiants et leur famille.

Le consensus est donc total : il n'y aura plus de tirage au sort, et le Gouvernement veillera à garantir la transparence du nouveau système d'accès à l'enseignement supérieur en y réintroduisant une part d'humain. largement, la problématique du premier cycle ne saurait se limiter à la question d'APB. Je rappelle que deux tiers des étudiants échouent à obtenir leur licence en trois ans. Nous devons à nos étudiants d'édifier un premier cycle qui leur permette de construire leur réussite plutôt que d'intérioriser dès le plus jeune âge l'échec comme horizon indépassable de leurs efforts. À cette fin, j'ai lancé le 17 juillet dernier une concertation sociale avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, afin de déterminer le contenu d'une réforme systémique du premier cycle. Tous les acteurs ont été entendus : établissements et représentants des étudiants, des élèves et de leurs parents. Nous prendrons prochainement une initiative législative globale sur le fondement du rapport final du recteur Daniel Filâtre qui m'a été remis le 19 octobre dernier, à l'issue de la concertation et des consultations que je conduis actuellement auprès des différents représentants de la communauté de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante. Cette réforme, qui sera globale, globale, permettra d'améliorer la réussite des étudiants. Je puis d'ores et déjà vous annoncer que nous garantirons la transparence du nouveau système en confiant sa gestion à un service à compétence nationale

remercie, madame la ministre, de votre réponse. Nous avons un certain nombre de convergences. Vous avez engagé une réflexion, mais je pense qu'il est maintenant temps de changer de système. Je souhaite vivement la mise en place d'une orientation bien en amont, qui tienne compte des aptitudes et des souhaits des futurs étudiants, mais aussi et surtout l'instauration de prérequis obligatoires à l'entrée de chaque filière.

L'impossibilité de retrouver les héritiers ou le refus des légataires d'accepter certaines successions immobilières au regard du mauvais état des bâtiments font que de plus en plus de communes sont affectées par des biens non entretenus, souvent au coeur même de leur centre-bourg. Ces biens se détériorant inexorablement jusqu'à devenir dangereux pour la population, les maires sont conduits à prendre des arrêtés de péril avant de devoir les faire démolir aux frais de leur commune. En effet, les domaines, qui,, deviennent propriétaires de ces biens « sans maître », répondent, lorsqu'ils sont sollicités par les élus, qu'ils ne disposent pas de ligne budgétaire à affecter à ces démolitions Ainsi les communes se retrouvent-elles seules à assumer indûment des travaux qui viennent grever des finances locales déjà fortement pénalisées par les baisses de dotation. À

qui, avec 2 000 habitants et un budget communal de l'ordre de 2 millions d'euros, va devoir financer dans les semaines qui viennent la démolition d'un bâtiment en centre-bourg pour un coût de 100 000 euros au minimum, d'autres cas similaires se profilant à brève échéance.

et suivants du code général des collectivités territoriales : après une procédure de constat d'un bien non entretenu et un échange avec le propriétaire, elle aboutit à une expropriation simplifiée pour cause d'utilité publique avec versement d'une indemnité.

En effet, à la suite de votre communiqué de presse du 27 septembre dernier, dans lequel vous avez fixé les orientations de la stratégie d'aménagement numérique des territoires, vous vous engagez à mobiliser l'ensemble des technologies disponibles, dont les solutions satellitaires nouvelles déployées, pour garantir à l'ensemble des foyers un accès au bon débit, c'est-à-dire entre 8 et 30 mégabits par seconde. Ce mixtechnologique est une bonne nouvelle. Comme nous le savons, des progrès industriels considérables ont pu être accomplis dans le domaine des télécommunications par satellite ces dernières années.

large échelle. Toutefois, la technologie satellitaire disponible à l'heure actuelle se heurte à un problème de saturation prégnant. Or les collectivités territoriales engagées dans l'aménagement numérique de leur territoire ont besoin de visibilité sur la part des foyers que cette technologie pourrait effectivement permettre d'atteindre,

dans quelle mesure le Gouvernement souhaite recourir à cette technologie, mais aussi comment les mesures de politiques publiques pourront faciliter la pénétration de cette solution en zone rurale au bénéfice des citoyens et des entreprises ? La parole

haut débit en 2020. Ce travail, réalisé en coordination avec les collectivités territoriales porteuses de projets de réseaux d'initiative publique, sera généralisé d'ici à la fin de l'année à l'ensemble des territoires.

la question n° 071, adressée à M. le ministre de la cohésion des territoires. Rabotage des aides personnalisées au logement, APL, baisse des loyers, exclusion des territoires ruraux du prêt à taux zéro et des bénéfices de la loi Pinel, et j'en passe ... Monsieur le ministre, toutes ces mesures inscrites dans le projet de loi de finances pour 2018 mettent à mal les territoires ruraux

moins tendues ? Tout simplement parce que, une nouvelle fois, on concentre l'avantage fiscal, et donc les investissements immobiliers locatifs, dans les territoires déjà urbanisés. Vous réservez les avantages fiscaux aux grandes villes et vous laissez mourir les milliers de zones qui ne sont pas des métropoles vous n'incitez pas les investisseurs à implanter leurs projets dans ces territoires plus reculés et plus fragiles économiquement. Ce sont pourtant ces zones qu'il faut soutenir pour favoriser leur développement ! En les excluant des avantages fiscaux, on les fait perdre en attractivité et on les fragilise encore davantage.

Les opérations neuves et de réhabilitation non lancées ne verront pas le jour et les actions sur le patrimoine, notamment en faveur de la qualité énergétique, seront dégradées. Il faudra alors expliquer aux locataires que, en contrepartie de la mesure populaire de baisse des APL, c'est la dégradation programmée de l'ensemble du parc social que vous allez mettre en marche c'est le retour vers le logement bas de gamme dans les secteurs détendus tels que le mien ... Je note enfin la brutalité de vos annonces, qui mettent à mal tout un écosystème, du bailleur social aux entreprises du BTP en passant par les architectes, les bureaux d'études, les promoteurs, les lotisseurs et les constructeurs.

pouvez-vous m'indiquer le montant des économies réalisées par le biais de ces mesures, mais aussi, et surtout, celui des pertes qui résulteront de l'abandon de ces dispositifs ? Le bilan ne risque pas d'être à l'avantage de nos finances publiques

de l'absence de baisse de dotation ni de la conservation au plus haut niveau des dispositifs de dotation et de subvention pour les communes. Toujours est-il que le bon sens, monsieur le sénateur, c'est d'avoir une approche équilibrée et juste de ce qui est fait.

Monsieur le ministre, ma question concerne des problématiques de politique éducative en milieu rural. Dans les départements qui connaissent une déprise démographique, les établissements du second degré perdent chaque année des élèves, et leurs internats se vident. internats se vident. Ainsi, dans les collèges du Cantal, il y avait, à la rentrée 2016, 128 internes ; il n'y en avait plus que 101 à la rentrée 2017, pour environ 600 places disponibles, dont près de 300 rénovées récemment. La possibilité de mettre en place des « internats liberté » a été évoquée. Comment cette mise en place est-elle envisagée ? Ces internats seront-ils proches des internats de la réussite pour tous, c'est-à-dire des internats que les jeunes choisissent pour les activités spécifiques qui y sont proposées ? Quel appui les collectivités territoriales peuvent-elles apporter à cette mise en place ? Les départements qui font face à des baisses d'effectifs préoccupantes dans leurs établissements du second degré pourraient-ils être prioritaires pour cette expérimentation ? La seconde partie de ma question concerne les regroupements pédagogiques intercommunaux, ou réseaux d'écoles de territoire. Lorsque la densité des effectifs est trop faible, les élèves, parfois de très jeunes enfants, sont confrontés à des temps de parcours très longs, particulièrement en zone de montagne. Est-il envisageable que ces territoires puissent bénéficier de mesures dérogatoires afin d'éviter des fermetures d'écoles qui imposeraient des temps de trajet excessifs ? La parole est à M. le ministre de la cohésion des territoires.

Lors de l'ouverture de la Conférence nationale des territoires, le 17 juillet dernier, au Sénat, le Président de la République a clairement marqué l'attachement du Gouvernement au service public de l'éducation dans les territoires ruraux.

entre l'État et les acteurs locaux à travers les conventions ruralité, pour que la totalité des territoires éligibles soient couverts d'ici à la fin de 2018.

concerne le collège et le lycée, le ministre de l'éducation nationale souhaite relancer le plan Internat en milieu rural, ce qui correspond à votre question. Actuellement, 200 000 lits sont disponibles en France, mais 20 % sont inoccupés, notamment en milieu rural. Revitaliser les internats ruraux à partir de projets d'excellence au sein des collèges et lycées rendus attractifs est de nature à donner une image positive de ces établissements, qui pourront devenir des lieux de réussite pour les élèves. Par ailleurs, le ministre de l'éducation nationale souhaite lancer une réflexion sur le rapprochement de l'école et du collège dans la ruralité, sur le plan tant du bâti que pédagogique.

Les structures chargées du dépistage précoce de l'autisme, les centres de ressources autisme, ou CRA, ont fait l'objet de virulentes critiques dans un récent rapport de Insuffisamment déployés sur le territoire national, parfois composés de personnes insuffisamment formées, surchargés au point de rendre leurs conclusions après des délais d'attente de près d'un an et demi, ces centres peinent à remplir leur mission. Le troisième plan Autisme avait fait de la réorganisation du réseau des CRA et de l'homogénéisation de leurs pratiques une priorité. Un décret du 5 mai 2017 a posé quelques « conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement Mais est-ce bien suffisant ? Peut-on se contenter d'un seul CRA par région ? Peut-on se satisfaire qu'un CRA doive parfois s'associer à un centre hospitalier spécialisé, autrement dit un hôpital psychiatrique, pour exister ? Comment peut-on tolérer que les recommandations de bonne pratique dont les CRA doivent se faire le relais ne soient nulle part mentionnées ? Les personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique se trouvent davantage exposées aux ruptures de parcours, aux carences de l'offre médico-sociale, à l'inadaptation des solutions actuellement proposées.

particulièrement, l'autisme. Les centres de ressources autisme ont été généralisés depuis plus de dix ans. Ils sont effectivement des acteurs majeurs dans le dispositif de prise en charge et d'accompagnement des personnes avec autisme. Vous indiquez que le récent décret régissant leur fonctionnement a été établi en 2017, sans concertation avec les usagers. Je veux vous rassurer : la publication tardive de ce décret, est travaillé depuis 2014, tient précisément à la durée des concertations et à la difficulté à trouver un point d'accord entre les nombreuses parties prenantes, comme trop souvent dans ce domaine, traversé par des débats et des conflits « plus délétères que féconds », selon l'expression du rapport d'évaluation du troisième plan Autisme. En l'espèce, il aura donc fallu trois ans pour confirmer, dans le décret de 2017, la place et le rôle central des CRA dans la chaîne repérage, diagnostic et intervention. Non pas toute la place, mais une juste place en tant que centre expert, pour les diagnostics les plus complexes, et centre ressources, pour la formation des équipes de proximité. une place essentielle pour garantir la fluidité d'un triptyque indispensable à la qualité des prises en charge, conformément aux bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé,

Je veux le dire clairement, la concentration des diagnostics sur les centres régionaux de ressources autisme est un vrai problème. Elle témoigne de l'insuffisance de la structuration des parcours et, surtout, de celle des outils donnés aux professionnels de santé et aux familles pour assurer une orientation adéquate.

Je sais compter sur l'engagement en ce sens de la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, qui est pleinement mobilisée sur le sujet, dans le cadre d'une feuille de route totalement croisée. La parole

la secrétaire d'État, la protonthérapie est une technique de radiothérapie utilisant des faisceaux de protons. Elle est aujourd'hui reconnue comme la méthode permettant de cibler le mieux une tumeur, tout en épargnant les tissus sains voisins. Moins toxique que la radiothérapie classique, elle permet notamment de s'attaquer à des cancers développés par l'enfant, tels que des tumeurs neurologiques ou de la colonne vertébrale. Chez l'adulte, ses bénéfices sont indiscutables dans le traitement des cancers de la prostate et des sinus. Le troisième plan Cancer, qui court sur la période 2014-2019, a prévu la création de nouvelles autorisations pour l'ouverture de centres de protonthérapie.

compte déjà plus de 760 000 habitants et jouit d'une situation géographique qui lui permettrait de répondre de la meilleure des façons aux enjeux d'égalité territoriale d'accès à ce traitement innovant, et ce, sur le plan aussi bien national que continental, du fait notamment de sa proximité avec la péninsule ibérique. De plus, forte de l'Oncopole, pôle de recherche sur le cancer et l'innovation en santé de dimension européenne, la métropole toulousaine peut déjà compter sur une dynamique médicale et scientifique de très haut niveau. Mobilisés depuis plus de trois ans sur ce dossier, médecins, chercheurs, ingénieurs, industriels et collectivités territoriales, solidairement rassemblés au sein du projet « protonthérapie et recherche Ils n'attendent plus aujourd'hui qu'un signe du Gouvernement pour engager les investissements qu'ils ont provisionnés. Aussi, madame la secrétaire d'État, pouvez-vous dès à présent nous préciser le calendrier, ainsi que les modalités pratiques de l'appel à projets de création de ces nouveaux centres de protonthérapie ?

L'accompagnement des évolutions technologiques et thérapeutiques, ainsi que le déploiement équitable de l'innovation en cancérologie figurent parmi les priorités de la politique menée par le Gouvernement. J'attire votre attention sur le fait qu'aucun appel à projets pour l'implantation de centre de protonthérapie n'est prévu par le plan Cancer 2014-2019. Dans le cadre de ce plan Cancer, l'Institut national du cancer, l'INCa, a remis au ministère de la santé son premier rapport sur le développement de la protonthérapie en juillet 2015. Il a mené des travaux complémentaires, en 2016, pour affiner les indications « projetées ». Se pose dorénavant la question de l'évaluation médico-économique de la protonthérapie, pour laquelle la Haute Autorité de santé doit être saisie. Cette évaluation permettra d'élaborer d'éventuelles recommandations de bonnes pratiques. Dans cette attente, les agences régionales de santé, les ARS, ont sursis à toute décision d'autorisation en la matière. Nous ne pouvons que souligner le mérite du positionnement volontariste du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de l'institut Claudius Regaud. Dans l'attente des orientations nationales, nous invitons ce projet à s'inscrire à moyen terme dans le cadre du processus d'autorisation

lequel sera mené en étroite collaboration et coordination avec le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. La parole de protonthérapie. Je regrette ce qui ressemble à un renoncement, bien qu'un engagement de l'État ait pourtant été acté sur ce sujet particulier de santé publique et de lutte contre le cancer. Nous pouvions espérer une autre réponse et une réelle volonté politique. La

Lorsqu'il ne conduit pas au décès, l'AVC constitue la première cause de handicap physique acquis chez l'adulte. Son coût pour l'assurance maladie est par ailleurs estimé à 4,5 milliards d'euros par an.

Face à ce phénomène, de nouvelles modalités de prise en charge ont été développées. Outre les traitements médicamenteux, la thrombectomie mécanique représente une avancée médicale capitale, permettant d'augmenter sensiblement les chances de survie des patients et de limiter les risques de séquelles. Encore faut-il que cette technique puisse être disponible sur tout notre territoire Si aujourd'hui ces traitements de pointe se développent au sein des unités neuro-vasculaires, unités spécifiquement dédiées à la prise en charge des personnes victimes ou suspectées d'AVC, de nombreuses zones géographiques, en particulier rurales, restent encore trop éloignées de ces structures, avec des temps de transport et d'acheminement bien trop longs. Or le délai de prise en charge d'un AVC est fondamental. On estime qu'une minute perdue représente en moyenne deux millions de neurones en moins ! Il est donc urgent d'assurer à nos

sont caractérisées par une incidence stable de 150 000 cas par an, avec un taux d'incidence multiplié par deux après 55 ans. La mise en oeuvre du plan AVC 2010-2014 a assuré non non seulement une restructuration de la prise en charge de la population au sein de filières AVC, mais aussi le développement d'outils d'aide à la décision pour réduire les délais de prise en charge. Je pense notamment à la télémédecine, avec la téléconsultation, la téléexpertise et la télésurveillance des AVC. L'innovation thérapeutique que représente la pratique de la thrombectomie mécanique par voie endovasculaire, couplée ou non à la thrombolyse, a montré une récupération quasi totale à trois mois, chez les personnes victimes d'infarctus cérébral, réduisant considérablement les risques de décès et de séquelles.

Elles sont proposées par le comité Thrombectomie créé à cet effet en février 2016, et qui réunit l'ensemble des acteurs impliqués, en lien avec les associations de malades France AVC et la Fédération nationale des aphasiques de France, la FNAF.

Le déploiement de cette activité s'inscrit également dans le calendrier de la réforme du régime des autorisations d'activités de soins, et de celui du troisième cycle des études médicales. Il repose aussi sur la télémédecine concernant les AVC, ou téléAVC, qui est l'un des éléments clés du parcours de soins. Plus de 30 projets de téléAVC sont inscrits dans les projets régionaux de santé, les PRS. À ce jour, une montée en charge progressive de l'activité est observée, notamment par un rattrapage dans les territoires sous-dotés en UNV et le travail se poursuit, avec l'ensemble des acteurs et avec un objectif fixé d'égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire.

des maladies cardio-vasculaires et cérébro-vasculaires qui permet d'impliquer tous les acteurs de la communauté médicale, mais aussi

n'envisage pas de mesures coercitives afin d'inciter fortement les médecins à s'installer dans les zones déficitaires. Il ne prévoit ni d'augmenter le des étudiants en médecine ni même de le supprimer. Or les pouvoirs publics vont être confrontés aux défis liés à la couverture médicale de l'ensemble du territoire, plus particulièrement dans les zones rurales et urbaines précarisées. Ce phénomène de désertification médicale est sans nul doute le résultat d'une conjonction de divers facteurs : un vieillissement des praticiens en activité, un recul des vocations de médecin généraliste, mais également un moindre attrait de l'exercice libéral. Ces réalités aboutissent à des situations extrêmement difficiles à gérer, telles des fermetures définitives de cabinets médicaux ou encore de maisons de santé « coquilles vides », entravant l'accès aux soins de nombreuses populations. Je voudrais citer pour exemple la ville de Huningue, dans le Haut-Rhin, comptant 7 000 habitants. Elle se voit privée de médecin généraliste depuis le 1 avril dernier, alors alors que, dès 2011, l'équipe municipale avait entrepris la création d'un pôle médical au coeur même de la commune, afin de pérenniser la présence des médecins généralistes. La municipalité s'est toujours montrée très attentive à l'ensemble des requêtes de ces professionnels de santé, tant en matière d'aménagement des locaux- des locaux fabuleux -que sur le calcul équitable des loyers et charges. Mais rien n'y a fait ! La situation est aujourd'hui inacceptable pour les élus locaux ! En réaction, les deux pharmaciens de Huningue ont lancé une pétition afin d'alerter les pouvoirs publics sur la pénurie de médecins.

qui pourraient figurer dans une réelle et ambitieuse réforme ! Partageant pleinement les légitimes inquiétudes exprimées tant par les patients que par les élus locaux sur ce sujet,

La réponse ne passe pas uniquement par la présence d'un médecin dans chaque village. Tout l'objectif du plan qui a été présenté par le Premier ministre et par Mme Agnès Buzyn est précisément d'ouvrir le champ des possibles en matière d'organisation, afin que les acteurs de terrain puissent mettre en oeuvre les solutions les plus adaptées à leur situation. Mme la ministre des solidarités et de la santé ne croit effectivement pas en la coercition ou au conventionnement sélectif. Cette méthode n'a pas démontré sa pertinence dans tous les pays qui l'ont essayée, car il y a toujours des moyens de contourner l'obligation. En outre, il semble essentiel de construire les réponses avec les professionnels, et non contre eux. sont prêts à prendre leur part de responsabilité, dès lors que nous leur facilitons la tâche en levant les verrous réglementaires. Aussi, ce plan est pragmatique et présente un panel de mesures destinées aux professionnels de santé et aux acteurs de terrain. Il s'inscrit autour de quatre objectifs importants redonner du temps médical au soignant, en facilitant les remplacements, le cumul entre emploi et retraite ou les exercices partagés entre ville et hôpital ; mettre en place la révolution numérique, en généralisant la télémédecine dès 2018 et en équipant toutes les zones sous-denses et les établissements coordonner les professionnels de santé entre eux, en doublant les maisons et centres de santé d'ici à cinq ans, notamment grâce au 400 millions d'euros d'aide à l'investissement issus du Grand Plan d'investissement

aujourd'hui, retardent l'âge de la maternité. Or, après 35 ans, il est scientifiquement démontré que la fertilité baisse. Le nombre d'ovocytes que peut produire une femme diminue progressivement, ce qui réduit ses chances lors de démarches de PMA, singulièrement pour

avec plus de 130 de ses confrères. Ils y affirment avoir aidé et accompagné des couples et des femmes célibataires dans leur projet d'enfant, dont la réalisation n'était pas possible en France. Ces mêmes professionnels se sont récemment émus de l'absence de positionnement favorable à l'autoconservation ovocytaire. Ainsi, de nombreuses Françaises vont bénéficier d'un diagnostic génétique embryonnaire ou d'une autoconservation ovocytaire

par les organismes représentatifs, à des établissements de santé privés ou publics, contrôlés par les pouvoirs publics. Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, de bien vouloir me donner votre avis, et par là même celui du Gouvernement, sur cette suggestion. La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, des personnes handicapées. L'extension de l'assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes relève de la loi. Elle mérite un débat apaisé. À l'heure actuelle, la PMA répond aux problèmes d'infertilité des couples hétérosexuels. Or les demandes d'accès à la PMA ont désormais vocation à répondre à d'autres problèmes. L'homoparentalité et la monoparentalité issues de cette technique sont, dans notre pays, une réalité. Chaque année- des chiffres ont déjà été cités -, 2 000 à 3 000 femmes ont légalement recours à la PMA dans des pays limitrophes. L'opinion publique évolue, puisque 61 % des Français sont favorables au recours à cette technique par les couples de femmes, alors qu'ils n'étaient que 55 % en 2014. Le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, a rendu un avis favorable à cette extension, le 15 juin dernier, en demandant de définir des « conditions d'accès et de faisabilité précisément de l'accès à l'insémination artificielle avec donneur aux femmes seules et aux couples de femmes. L'avis va vers plus d'autonomie pour les femmes, conforté par l'absence de violence engendrée par cette technique et par la relation à l'enfant, satisfaisante, dans ces nouvelles structures familiales. Le CCNE s'inquiète d'un maintien du, qui stigmatiserait ces formes familiales. Cependant, il recommande des conditions d'accès et de faisabilité pour les femmes seules, plus vulnérables, ainsi qu'une gratuité garantie du don de gamètes. Vous le savez, l'actuelle loi de bioéthique du 7 juillet 2011 sera révisée l'an prochain. Conformément aux dispositions prévues, cette révision sera précédée de la tenue d'états généraux, sur l'initiative du CCNE. Le sujet de l'extension de la PMA pourra être débattu, au premier semestre 2018, lors de ces états généraux. Ce n'est qu'ensuite que sera élaboré le projet de loi de bioéthique. Il est donc trop tôt pour connaître les dispositions qui seront contenues dans ce projet de loi. La parole

une analyse chromosomique est autorisée en France pour les femmes enceintes qui le souhaitent, pour un dépistage anténatal, mais cela reste interdit pour le prélèvement d'une cellule sur l'embryon, avant le transfert, ce qui nous paraît incohérent. La

Chaînons essentiels de notre industrie laitière, mais également protecteurs indispensables de la santé de nos concitoyens, les laboratoires d'analyse de lait ne bénéficient pourtant pas du même régime que les laiteries concernant le travail dominical. Contrairement à ces dernières, qui profitent en permanence d'une dérogation au titre des denrées périssables, les laboratoires d'analyse de lait, acteurs essentiels de la santé publique, ont besoin d'une dérogation renouvelable annuellement pour pouvoir travailler le dimanche. Le laboratoire d'analyse MyLab, reconnu par les pouvoirs publics, situé sur ma commune de Châteaugiron, en Ille-et-Vilaine, s'occupe de l'analyse laitière à destination de 65 laiteries et de près de 20 000 fermes dans la zone Grand Ouest. Il a ainsi attiré mon attention sur cette situation préoccupante. La dérogation demandée est essentielle pour trois des activités de ces laboratoires : la collecte des échantillons l'astreinte pour assurer la conformité à la réglementation sur le critère de résidus d'antibiotiques dans le lait ; l'astreinte pour assurer la surveillance vis-à-vis des critères bactériologiques. La demande annuelle d'une telle dérogation est donc un frein administratif au bon déroulement de l'activité à caractère sanitaire de ces structures. Les lourdeurs administratives peu pertinentes- voilà l'incongruité dont je parlais -telles que la nécessaire délibération du conseil municipal de la commune où se situe le laboratoire constituent un véritable problème pour ces laboratoires. C'est une difficulté importante et assez incompréhensible qui peut mettre en danger l'activité de ces acteurs de la santé publique.

La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées. Madame la sénatrice Gatel, je vous prie de bien vouloir excuser ma collègue Muriel Pénicaud, qui est retenue par les concertations avec les partenaires sociaux sur le deuxième volet de la transformation de notre modèle social. Vous interrogez le Gouvernement au sujet des conditions d'autorisation du travail dominical des laboratoires d'analyse de lait, plus précisément du laboratoire MyLab, situé à Châteaugiron. Comme vous l'indiquez, ces laboratoires d'analyse de lait ne bénéficient pas, contrairement aux laiteries qu'ils contrôlent, d'une dérogation permanente au repos dominical au titre du code du travail. Néanmoins, cette activité d'analyse peut bénéficier d'une dérogation au repos dominical au titre du code rural et de la pêche maritime. En effet, les articles L. 714-1 et R. 714-1 de ce code le permettent, sous réserve toutefois que les organismes de contrôle laitier

Dans ces conditions, en l'état actuel du droit et à moins d'une modification de son régime d'affiliation, le laboratoire MyLab doit continuer à solliciter auprès du préfet une dérogation temporaire au repos dominical, sur le fondement de l'article L. 3132-20 du code du travail. La parole

c'est quand même une curiosité française dont on pourrait se passer pour plus d'efficacité et de sécurité. La parole

Madame la secrétaire d'État, je veux attirer votre attention sur les conséquences inquiétantes de la diminution drastique et immédiate du nombre de contrats aidés dans nos communes et nos territoires. Je prends un exemple simple, celui de la commune d'Audincourt, ville de 15 000 habitants, qui, à travers ses associations, se voit profondément impactée par cette décision.

auxquels s'ajouteront trois autres contrats aidés au cours de la période 2017-2018. L'association Réussir Ensemble, située également aux Champs-Montants, s'est vu refuser le renouvellement de deux contrats aidés. L'association Soli-cités, une association d'aide et de soins à domicile, doit normalement renouveler douze contrats aidés d'ici à la fin de l'année, des emplois qui représentent un souffle indispensable pour cette structure. Les Francas du Doubs nous alertent également, tout comme nous fait part de ses plus vives inquiétudes puisque la perte et le remplacement par des agents des services hospitaliers des quinze contrats aidés que compte cette structure représentent un coût supplémentaire de 65 600 soit une augmentation du prix de journée de 4,35 euros. Voilà, madame la secrétaire d'État, à l'échelle d'une ville moyenne, un tableau rapide et non exhaustif des conséquences concrètes d'une telle décision. Diminuer drastiquement et sans aucune concertation le nombre d'emplois aidés a non seulement comme conséquence directe le retour à la précarité pour les personnes concernées, un coup porté à la cohésion sociale et aux services rendus aux plus fragiles qui sont directement remis en cause. Madame la secrétaire d'État, pouvons-nous avoir un débat sur ces questions, d'assurer le vivre ensemble dans les quartiers, éviter des drames et, certainement, une remise en cause durable de la cohésion sociale

Vous demandez au Gouvernement de maintenir l'ensemble des contrats aidés, alors que vous aviez non seulement sous-budgétisé ce dispositif- 280 000 contrats aidés en loi de finances initiale pour 2017 contre 459 000 en 2016 -, mais aussi consommé plus des deux tiers des crédits de l'enveloppe au premier semestre. Face à cette situation, et dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, le Gouvernement a pris ses responsabilités en accordant 40 000 contrats aidés de plus. Ceux-ci sont recentrés sur les publics les plus éloignés du marché du travail et là où ils sont indispensables à la cohésion sociale et territoriale, notamment en direction des communes rurales en difficulté financière extrême. Au-delà, nous considérons qu'une politique de l'emploi efficace, capable de répondre aux défis à venir, doit s'appuyer sur le renforcement des politiques de formation et d'accompagnement ciblé qui donnent plus d'atouts, de capacités aux personnes qui en bénéficient pour s'insérer durablement dans l'emploi. C'est le sens du Grand Plan d'investissement compétences, d'un montant de 15 milliards d'euros, de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, mais aussi de la mission que Muriel Pénicaud a confiée à Jean-Marc Borello, président du Groupe SOS, pour apporter des solutions d'insertion innovantes et accompagner également les associations pour une nouvelle gouvernance, ce qui leur permettrait de faire face à ces difficultés financières. je vous remercie elles n'ont pas ces contrats aidés ? Vous nous parlez de maîtrise des dépenses publiques ; il y a d'autres choix à faire. Vous avez supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, vous avez fait des choix.

de renouer le dialogue avec le Gouvernement et de revoir cette politique des contrats aidés, nous pourrions certainement entamer une vraie discussion et, surtout, essayer de sortir de cette situation.

dans le système scolaire, ils mènent des actions sociales indispensables : c'est la lutte contre l'échec scolaire. Tout cela va s'arrêter au mois d'octobre, au mois de novembre, si nous ne trouvons pas une solution. Parfois, Parfois, il faut entendre le bon sens. Ce n'est pas une intervention politique partisane que je fais aujourd'hui ; j'essaie d'attirer l'attention du Gouvernement sur un risque grave pour la cohésion sociale dans les quartiers.

mes chers collègues, la France est la première destination touristique mondiale, avec plus de 80 millions de visiteurs en France métropolitaine en 2015. Représentant 8 % du PIB et deux millions d'emplois directs et indirects, le tourisme est un secteur clé de l'économie française. Il ne serait pas bon de se reposer sur nos lauriers. Car, nous le savons, l'année 2016 a été très mauvaise en raison des attentats. Nous devons renforcer notre offre touristique et l'attractivité de la France. Les défis ne manquent pas, au premier rang desquels la sécurité, mais aussi le numérique avec l'e-commerce et le travail à domicile, le tourisme des seniors, le boom du tourisme chinois, une meilleure valorisation du patrimoine, le problème des coûts élevés, la piètre qualité de l'accueil des étrangers, etc. Nous devons aussi adopter des ajustements en matière de fiscalité pour promouvoir l'investissement, adopter des simplifications administratives. Je soulignerai deux autres points qui mériteraient l'attention et la vigilance du Gouvernement : d'une part, la question du renouvellement des clientèles, notamment l'adaptation de l'offre touristique aux besoins des jeunes générations d'autre part, la question centrale des transports, individuels et en commun. Ce point détermine la capacité de développement des stations. Concernant la destination Savoie-Mont-Blanc, territoire dynamique dont nous souhaitons développer les atouts « quatre

Il faudrait revenir également sur la législation concernant les unités touristiques nouvelles qui, trop complexe, pénalise les nouveaux projets en pays de Savoie. De plus, les normes françaises concernant l'hôtellerie familiale pénalisent lourdement la transmission et impliquent des fermetures nombreuses. Inspirons-nous de la Suisse et de l'Autriche. Concernant les modifications du calendrier scolaire pour une saison de ski plus longue, des efforts ont été faits, mais ils doivent être poursuivis. Monsieur le secrétaire d'État, quelles actions le Gouvernement compte-t-il entreprendre en faveur de ce secteur ? Pourriez-vous nous détailler la politique du tourisme qu'il souhaite mettre en oeuvre pour atteindre les 100 millions de touristes internationaux en 2020 ? La parole

Même si la conjoncture du tourisme se redresse en 2017, vous l'avez souligné dans votre propos, il ne faut pas oublier la contre-performance de 2016- baisse du nombre d'arrivées de touristes internationaux de 2,2 % -, consécutive aux attentats terribles terribles qui ont frappé l'Hexagone. Cela montre que la compétitivité du site France n'est jamais acquise et qu'il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, qu'il faut poursuivre les efforts qui ont été engagés, parfois depuis longtemps, au-delà des appartenances partisanes. La politique du Gouvernement a été définie lors du comité interministériel du tourisme qui s'est tenu à Matignon le 26 juillet dernier et dont les grandes orientations ont été rappelées il

Cela passe par la rapidité dans la délivrance des visas- des efforts ont été engagés en ce sens -et par la promotion de la marque d'État Qualité Tourisme. Deuxième axe

-, qui permettent de fédérer les acteurs d'un territoire autour d'une stratégie touristique commune de structuration et de promotion de l'offre touristique, afin de rendre l'offre de la destination France plus lisible. La politique des contrats de destination sera poursuivie en 2018 avec la continuation des premiers contrats qui arrivent à échéance. Troisième axe : le soutien étatique en matière d'investissements, qui suppose une meilleure mobilisation du fonds France Développement Tourisme, doté de 1 milliard d'euros sur cinq ans. Mis en place en 2015, il a permis de mobiliser des crédits de la Banque publique d'investissement et de la Caisse des dépôts sur les entreprises et projets touristiques porteurs. Le Gouvernement vient en outre de lancer une mission pour identifier les propositions qui permettront de faciliter la rénovation du parc privé d'hébergements touristiques, notamment dans les stations littorales et de montagne- ces dernières vous sont chères, monsieur le sénateur, et je connais bien, moi aussi, cette région de la Savoie dont vous êtes l'élu. Quatrième axe : la formation et l'emploi. Le Gouvernement a fait des formations dans le secteur du tourisme l'un des enjeux majeurs du développement du secteur. Il s'agira de poursuivre

dispensées par une douzaine d'établissements, ont été sélectionnées et l'appel à candidatures reste ouvert. Le Gouvernement souhaite également augmenter le nombre de contrats d'apprentissage dans le secteur, en concertation avec les professionnels, pour développer l'offre des entreprises en direction des moins de 25 ans et lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Le secteur touristique

Cinquième axe : le soutien à la numérisation et au partage d'informations. Cette action comprend le développement de DATAtourisme, évoqué dès le comité interministériel du 26 juillet dernier,

En tout cas, nous nous assurerons de la mise en oeuvre de ces axes dans le cadre des comités interministériels du tourisme et de leurs comités de pilotage, qui se réunissent tous les trois mois, et dont vous aurez bien évidemment connaissance. La parole

Monsieur le secrétaire d'État, ma question porte sur l'état d'avancement des discussions entre les services du ministère chargé du tourisme et les opérateurs présents en ligne référençant les activités touristiques. Depuis novembre 2016, à la suite de l'évolution des procédures utilisées par ces groupes puissants en situation de quasi-monopole, l'ensemble des offres touristiques présentes sur le territoire de plusieurs collectivités ne sont plus du tout référencées. De fait, un cloisonnement géographique a été mis en place. Par exemple, avant cette date, une recherche effectuée sur des sites comme TripAdvisor et Booking permettait d'associer au nom « Carcassonne » l'ensemble de l'offre touristique présente sur les communes avoisinantes. Depuis près d'un an, ce n'est plus le cas. À cause du cloisonnement géographique mis en place par ces référenceurs, même un établissement présent à moins d'un kilomètre de la cité médiévale, mais domicilié sur une autre commune que Carcassonne, ne se voit plus identifié dans les possibilités offertes aux clients. Même la communauté d'agglomération se trouve impactée puisqu'elle ne peut plus référencer ses offices du tourisme communautaires en les rattachant à la ville-centre. Vous en conviendrez, monsieur le secrétaire d'État, c'est fortement dommageable. À la suite de cette évolution, certaines activités touristiques ont subi une large baisse de fréquentation, allant jusqu'à près de 30 % dans le département de l'Aude. C'est d'autant plus pénalisant que des acteurs touristiques continuent de payer pour être référencés, certains ayant même choisi de s'appuyer principalement sur ces groupes pour assurer leur communication. Pourquoi une telle situation ? Il apparaît dans les échanges avec ces grands groupes qu'ils ont souhaité standardiser leurs procédures, mais qu'ils ont pris néanmoins conscience des limites de ces dernières, notamment au vu des multiples réclamations dont elles ont fait l'objet. en raison des enjeux pour les professionnels du tourisme et pour nos collectivités, j'aimerais connaître l'état d'avancement des discussions entre vos services et les grands opérateurs. Je souhaite sincèrement qu'une solution rapide et pérenne puisse être apportée.

par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en présence de plusieurs membres du Gouvernement et d'une trentaine de professionnels représentatifs des différentes activités touristiques. À l'occasion de cette réunion a été annoncé le lancement d'une mission sur le financement de la promotion de la destination France qui devra rendre ses conclusions avant la fin de l'année.

les grands acteurs numériques qui bénéficient de ses actions de promotion sans pour autant les financer- en tout cas pas toujours. L'Union nationale pour la promotion de la location de vacances, qui regroupe notamment les grands acteurs numériques tels que Airbnb, Abritel Homeway, Expedia et TripAdvisor, représentée par son président, a participé à ces travaux et redit sa volonté de contribuer à l'effort collectif selon des modalités qu'il appartiendra aux trois rapporteurs de la mission de définir. Sur la question plus spécifique du référencement des professionnels les services du ministère ont été saisis d'une situation préoccupante à Carcassonne, sur votre territoire. La plateforme TripAdvisor a en effet décidé de changer son découpage territorial

pas toujours des plus opérationnelles et efficaces, et fédérer les acteurs territoriaux du tourisme autour d'une marque commune. Le contrat de destination « Pays cathare » est d'ailleurs le reflet de cette ambition et il bénéficie à plein de ce dispositif. Après plusieurs échanges, TripAdvisor a indiqué avoir pris conscience des problèmes générés par son nouveau découpage territorial et travaille à des fonctionnalités moins restrictives pour les professionnels. La plateforme nous a indiqué traiter le cas de Carcassonne en priorité et doit faire des propositions dans le courant du mois de novembre. Elle est en relation constante avec l'office du tourisme du Grand Carcassonne et les services du Quai d'Orsay pour apporter au plus vite une solution satisfaisante à cette situation pour le moins ubuesque. Ce cas particulier de Carcassonne n'est pas isolé en France ; d'autres

pour la protection que la sécurité sociale offre à nos compatriotes et, même si cela est peut-être moins connu, pour la densité et le dynamisme de notre réseau diplomatique et consulaire. La France permet ainsi à ses ressortissants installés ou de passage à l'étranger de bénéficier d'un réseau en constante évolution et dont nous avons toujours préservé l'universalité. Aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'État, je souhaite vous interroger sur la façon dont votre ministère gère les personnels qui animent ce réseau. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères est un employeur atypique : il fait travailler près de 14 000 agents aux statuts très différents, dont un tiers d'agents de droit local. Cette catégorie de personnel regroupe des agents aux profils et aux fonctions très variés, recrutés localement par nos postes et soumis à la législation locale. À l'instar de leurs collègues titulaires, ils doivent en permanence s'adapter à des méthodes de travail qui se modernisent. Dans le même temps, sont aussi tenus de respecter le référentiel Marianne qui garantit un accueil efficace et courtois aux usagers dans nos consulats. Le contexte budgétaire a conduit le ministère, afin de faire des économies, à remplacer, sur certains postes, des agents titulaires par des recrutés locaux dont le traitement salarial est tout à fait différent. Au vu de la forte activité des postes, la contribution de ces agents à notre réseau diplomatique, consulaire et culturel est devenue à la fois incontournable et fondamentale. Or je suis inquiète de constater, au fil de mes déplacements, la dégradation des conditions de vie de ces agents. Les revalorisations salariales consenties par le ministère sont très insuffisantes au regard du coût de la vie dans les grandes villes comme Toronto, New York, San Francisco, ou encore Istanbul, dont je reviens, où leurs salaires ne sont plus en phase avec l'augmentation des loyers et des transports. Les recrutés locaux célibataires ou ayant une famille à charge ont de grandes difficultés à se loger décemment. Certaines situations individuelles sont tout à fait critiques. Monsieur le secrétaire d'État, je ne peux me résoudre à ce que des agents qui travaillent au service de la France depuis de nombreuses années ne puissent vivre dignement. Aussi, je voudrais connaître les mesures que vous comptez prendre pour répondre aux préoccupations pour répondre aux préoccupations de ces personnels et, en premier lieu, leur assurer à toutes et à tous des conditions de travail et de vie décentes. La parole

du Sud ou en Tunisie plus récemment avec le Premier ministre. Ces agents représentent 46 % des effectifs du ministère de l'Europe et des affaires étrangères à l'étranger. Ce ministère est évidemment très attentif à la situation de ces personnels dans l'ensemble du réseau, en particulier aux États-Unis, compte tenu du coût élevé de la vie en Amérique du Nord. Dans un contexte budgétaire contraint, il s'assure tous les ans que les conditions de rémunération de ces personnels sont adaptées à l'évolution du coût de la vie et à la politique salariale pratiquée chez nos principaux partenaires dans les pays considérés.

Ce point précis répondait à une préoccupation souvent exprimée par les personnels locaux. Par ailleurs, 22 pays verront leurs cadres salariaux révisés à compter du 1 janvier 2017, afin de les adapter aux conditions locales de rémunération, pour un coût annuel total de plus de 1,6 million d'euros. Ces montants illustrent l'effort budgétaire significatif consenti par le ministère en faveur des agents de droit local dont l'importance Les agents de droit local aux États-Unis ont pu bénéficier, au cours des dernières années, d'augmentations régulières et significatives. Ces revalorisations ont été mises en place sur plusieurs années consécutives. Sur la base d'une étude des niveaux de salaire offerts aux agents de droit local dans l'ensemble de nos postes aux États-Unis, une revalorisation vient d'être décidée, pour les villes où un décrochage est patent par rapport à nos partenaires européens. Une revalorisation uniforme de 2 % a été accordée aux agents à New York et à San Francisco. Le cas du Canada pourra être étudié de la même manière en 2018. Les agents de droit local aux États-Unis ont régulièrement bénéficié des augmentations annuelles au titre du mécanisme du coût-vie, sans préjudice des revalorisations structurelles que je viens de rappeler. En ce qui concerne l'accès aux concours internes de la fonction publique, le ministère étudie plusieurs pistes, à la fois juridiques et statutaires, qui permettraient aux agents de nationalité française d'accéder à des modes de recrutement ouvrant la voie à une intégration dans un corps du ministère. L'action de ces agents au quotidien est au quotidien est déterminante pour le bon fonctionnement de notre réseau diplomatique et consulaire. Enfin, s'agissant de l'éligibilité à l'indemnisation chômage des recrutés locaux qui rentrent en France, il est exact que le cadre juridique de ce mécanisme de protection ne permet pas d'en faire bénéficier les employés ayant exercé dans notre réseau sous contrat de travail de droit étranger et décidant de rentrer en France. Il s'agit d'un sujet sur lequel nous devrons nous pencher rapidement.

ont organisé des études comparatives entre les salaires que nous octroyons à nos recrutés locaux et les salaires versés par d'autres ambassades dans leur pays de résidence.

grand nombre de recrutés locaux quittent leur poste, tout simplement parce qu'ils perçoivent des salaires plus intéressants ailleurs, alors que nous avons vraiment besoin de ces personnels bilingues,

Normand. Historiquement, l'exploitation de la craie, aussi appelée marne, était utilisée pour enrichir la terre agricole. Les exploitations souterraines accessibles par un puits sont aujourd'hui de loin les plus nombreuses nombreuses en Normandie. En effet, les extractions de marne devaient se situer à proximité des surfaces agricoles situées sur les plateaux où la craie est en moyenne à 25 mètres de profondeur. Ces cavités étaient accessibles par un puits, qui permettait de descendre dans des galeries, créant une véritable toile d'araignée souterraine. En Seine-Maritime, le volume de chaque marnière vide était environ de 250 mètres cubes. Quand la marnière n'était plus exploitée, le puits était refermé et signalé par un arbre.

depuis plusieurs années, sous l'impulsion notamment de mon collègue le sénateur Charles Revet, la législation a évolué pour mieux prendre en compte le dommage résultant de l'effondrement des marnières. Dorénavant, l'état de catastrophe naturelle peut être reconnu sous certaines conditions et le Fonds Barnier permet de financer la prise en charge partielle des opérations de sondage et de comblement. à ces situations récurrentes, les maires jouent un rôle central, au titre tant de leur pouvoir de police, notamment par l'adoption d'un arrêté de péril ou la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, que du relogement des sinistrés.

dans mon département, l'Eure. L'exploitation passée des marnières, pour extraire de la craie dans le sous-sol, a duré des siècles dans notre région et provoque des effondrements, parfois terribles, vous l'avez rappelé.

Les travaux de prévention engendrent des coûts importants, qu'il n'est pas toujours évident de prendre en charge. Aussi, le Fonds Barnier s'applique pour les opérations de reconnaissance et les travaux de comblement ou de traitement des cavités souterraines, avec une subvention à hauteur de 30%, et pour les études et travaux de réduction de la vulnérabilité, prescrits dans le cadre d'un plan de prévention des risques, ou PPR, avec une subvention à hauteur de 40 % pour les habitations et de 20 % pour les biens à usage professionnel des petites entreprises.

Monsieur le secrétaire d'État, ma question porte sur la stratégie que le Gouvernement compte mettre en oeuvre concernant la présence du loup dans nos territoires et tout particulièrement le plan Loup 2018-2023. Pour que les troupeaux et les loups cohabitent, l'État a instauré un arsenal d'interventions telles que la dissuasion par effarouchement, le tir de défense ou le tir de prélèvement avec un quota annuel de loups qu'il est possible d'abattre. Une des caractéristiques du pastoralisme dans les Alpes-Maritimes est que les troupeaux restent en extérieur quasiment toute l'année, ce qui explique la raison en 2016, mon département a enregistré le plus d'attaques de troupeaux- près de 3 000 bêtes - et le plus de tirs de prélèvement- 14 -, selon un décompte de la Compte tenu de cette particularité, le quota de loups abattables est de 42 jusqu'au 1 janvier 2018, mais déjà, à l'heure actuelle, 29 loups ont dû être abattus contre 30 à Noël dernier. Ce plafond sera donc vraisemblablement dépassé. Le ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a déclaré qu'il souhaitait rencontrer toutes les parties prenantes après l'été 2017, afin de pouvoir définir une stratégie claire pour les prochaines années. Mais la situation est urgente, les éleveurs sont inquiets face aux premières propositions du plan Loup 2018-2023, qui ne prend pas en compte leur première préoccupation : mieux protéger leurs troupeaux. La problématique n'est pas spécifique aux Alpes-Maritimes,

Pouvez-vous présenter la méthode que le Gouvernement compte employer pour remettre les éleveurs au coeur du dispositif, pour la sauvegarde des activités pastorales et rurales ? Alors même que la première réunion nationale sur le loup organisée le 22 juin 2017 à Lyon n'a pas été très concluante et qu'une première manifestation d'éleveurs s'est déroulée récemment contre les premières mesures proposées dans le plan Loup, le Gouvernement compte-t-il amender son plan d'action et écouter les éleveurs ? Enfin, les collectivités locales auront-elles un rôle spécifique dans les territoires concernés par ce plan quinquennal ? La parole

ne partons pas de zéro. Les différents plans nationaux Loup ont permis la mise en place de mesures indispensables pour financer les moyens de protection des troupeaux, vous l'avez rappelé, indemniser les éleveurs, mais aussi assurer un dialogue entre les différents acteurs.

pour assurer la défense des troupeaux tout au long de l'année 2017, notamment dans votre département, madame la sénatrice. Quel est l'objectif visé par le Gouvernement ? Nous voulons aboutir à l'élaboration du prochain plan Loup dès 2018, dont le principal enjeu sera de garantir la viabilité de l'espèce sur le territoire- c'est une nécessité -, tout en contribuant à réduire considérablement la prédation des troupeaux. Cet objectif est bien évidemment partagé par le ministre de l'agriculture et le ministre de la transition écologique. Quelle est la méthode du Gouvernement ? Nicolas Hulot a décidé de remettre à plat

du pastoralisme confronté aux prédations. Là aussi, des perspectives d'amélioration sont à noter. Je citerai encore les foyers d'attaque ou l'impact des tirs sur la régulation de la prédation et sur la démographie de l'espèce. Sachez que, dans le cadre de ce prochain plan, les collectivités territoriales seront appelées à apporter leurs compétences et leurs moyens pour mettre en oeuvre plusieurs actions. Je pense notamment à l'accompagnement des éleveurs et à l'amélioration des conditions de vie pastorale. C'est ainsi que l'ont formulé les acteurs locaux lors de déplacements ministériels. Ils souhaitent intervenir dans un

Quelles sont les clés de lecture qui permettraient aux collectivités locales de prendre des décisions pertinentes sur le long terme ? dans le cadre de l'application de la loi dite de transition énergétique. Nous savons que la valorisation matière des déchets doit atteindre 65 % à l'horizon de 2025 et que l'enfouissement des déchets doit être réduit de 50 à la même échéance. Les collectivités intègrent la nécessité d'agir à la source en accordant la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets pour parvenir à l'objectif de réduction de 10 % des quantités de déchets en 2020 par rapport à 2010. Partout en France, monsieur le secrétaire d'État, des réflexions sont conduites pour adapter les unités de traitement de nos territoires et répondre à nos enjeux. Les investissements à prévoir engagent l'avenir de nos concitoyens qui assument le coût du service de collecte et de traitement des déchets au travers de la taxe ou de la redevance dédiée. Il importe, pour faire les choix technologiques les plus performants, que le Gouvernement donne ses intentions, sa position. Dans un avis de mars 2017 intitulé, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, semble faire la part belle aux usines d'incinération. Je ne comprends pas, monsieur le secrétaire d'État, que les réticences soient aussi fortes envers les unités de prétraitement des ordures ménagères, alors qu'il s'agit d'installations capables de valoriser de 50 % à 90 % des ordures ménagères entrantes. Plusieurs opérateurs sont en mesure aujourd'hui de proposer des unités s'appuyant sur les technologies existantes et en prenant partie de produire du combustible solide de récupération, CSR, ou d'utiliser la méthanisation. Il me semble que l'esprit de la loi de transition énergétique est d'encourager les initiatives innovantes plutôt que de les limiter. Exactement ! Je vous demande également de nous éclairer sur la trajectoire de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP. TGAP. Prévoyez-vous de l'augmenter dans les années à venir ? À quel rythme ? Pouvez-vous nous donner des objectifs chiffrés qui permettront ainsi aux collectivités d'apprécier la conduite à tenir ? Technologie, innovation, trajectoire financière : quelle est la visibilité pour nous permettre de prendre des décisions pertinentes ?

minutes trente pour la stratégie sur les déchets, c'est court ! Je vais tenter d'être concis et efficace. Quels sont nos objectifs ? C'est la continuité de la loi que le Parlement a a votée sur la transition énergétique, comme la continuité dans la volonté de diminuer nos gaz à effet de serre. Vous savez à quel point la question du recyclage permet d'y parvenir. C'est l'un des axes forts du plan Climat qui a été dévoilé par Nicolas Hulot, vous le savez, au mois de juillet dernier. dernier. Au moment même où nous nous parlons dans cet hémicycle, monsieur le sénateur, Brune Poirson est en train de présenter la méthode qui permettra l'élaboration de la feuille de route sur l'économie circulaire, afin de lancer une grande période de concertation avec l'ensemble des acteurs, y compris les élus locaux très fortement engagés dans les syndicats de traitement des ordures ménagères pour lesquels nous devons avoir le plus grand respect et la plus grande écoute. Comment allons-nous atteindre les objectifs ? C'est la vraie question, monsieur le sénateur. Tout d'abord, nous devons beaucoup progresser dans notre pays, vous l'avez dit, en termes de déploiement du tri des déchets. C'est un enjeu majeur. Sur ce sujet, les intentions du Gouvernement sont claires, notamment sur la trajectoire prévue de la TGAP. Conformément à l'engagement du Président de la République pendant sa campagne, nous augmenterons cette taxe collectée sur la mise en décharge et l'incinération d'ici à la fin du quinquennat. C'est là une condition indispensable Pour rendre le recyclage plus compétitif que la mise en décharge, il faut créer l'effet de levier. Nous le savons, il est néanmoins nécessaire que cette évolution soit soutenable pour les entreprises et les collectivités territoriales. Cela signifie deux choses : d'une part, monsieur le sénateur, les augmentations ne doivent pas avoir lieu trop tôt, pour laisser le temps

ne permettent généralement pas la production d'un compost de qualité pure : les composts produits contiennent encore, notamment, des morceaux de plastique. C'est pourquoi la loi privilégie explicitement la mise en place du tri à la source des biodéchets et indique, dans ce cadre,

développement d'installations innovantes, à la seule condition qu'elles soient compatibles avec le déploiement du tri à la source, qui est nécessaire pour assurer un recyclage ou un compostage de qualité. Ces questions très techniques

On ne peut donc se tromper ni sur les choix financiers ni sur les choix techniques. Nous comprenons bien que le Gouvernement veuille assurer la continuité de l'application de la loi- il n'y a pas de débat sur

de l'utilisation de techniques telles que la méthanisation ? Quelle est la part d'innovation que vous nous laissez ? Vous venez aussi de m'indiquer que

nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Tours-Bordeaux. Depuis le 2 juillet 2017, date de mise en service de cette ligne, les riverains immédiats mais aussi, parfois, les résidents de villages distants de la ligne ressentent les nuisances sonores ou vibratoires occasionnées par

à l'échelle de l'ensemble de la ligne que sur les sites les plus sensibles, conformément aux normes en vigueur pour une telle situation, en particulier l'arrêté du 8 novembre 1999. La réglementation prévoit que les mesures réalisées prennent en considération le niveau sonore moyen sur deux périodes de référence. Les pics de bruit, qui sont en réalité ce qui affecte le plus les riverains, ne comptent pas aujourd'hui parmi les mesures retenues. LISEA a également indiqué privilégier, dans sa sélection

au-delà de cette limite, notamment les hôpitaux, les écoles et les sites qui accueillent un public sensible, afin d'y prendre en considération les pics de bruit répétés au cours de la journée. Ces deux points révèlent que le respect de la réglementation en vigueur, sur laquelle LISEA entend se fonder pour réaliser les infrastructures de protection acoustique des riverains, risque de ne pas suffire pour protéger pleinement ceux-ci des nuisances. J'entends dès lors interroger par votre intermédiaire, monsieur le secrétaire d'État, Mme la ministre chargée des transports quant aux possibilités, d'une part, de prendre des mesures de protection complémentaires à celles existant aujourd'hui et, d'autre part, de faire évoluer la réglementation applicable afin d'apporter une

riverains de la nouvelle infrastructure, qui s'inquiètent des nuisances sonores occasionnées. Le Gouvernement a pleinement conscience de ce problème. Nous avons été saisis directement par des associations d'élus et des parlementaires ; vous le faites encore ce matin, madame la sénatrice. Quel est le cadre prévu pour ces nuisances sonores ? Les impacts sonores des nouvelles infrastructures de transport sont strictement encadrés par la réglementation. Je veux ici vous confirmer que le concessionnaire, LISEA, devra scrupuleusement respecter les niveaux maximums

a demandé aux préfets concernés d'organiser des comités de suivi, qui associent la population, pour veiller au respect de la réglementation par LISEA, mais surtout pour recenser les difficultés apparues et les faire remonter au ministère, ce qui nous permettra d'avoir un dialogue opérationnel et concret avec le concessionnaire.

favorable à ce que le Fonds de solidarité territoriale de la LGV Sud-Europe-Atlantique soit mobilisé pour toute action visant à améliorer l'insertion environnementale de la nouvelle infrastructure

Dans ce cas, et sous la présidence du préfet coordinateur, un financement pourrait être mis en place. Mme Élisabeth Borne aura en tout cas à coeur de réunir les collectivités territoriales concernées dès le début de l'année 2018, partant du résultat des mesures

qui roulent entre Paris et Bordeaux et qui ont été utilisées par LISEA dans le cadre des prémesures acoustiques avant l'ouverture de la ligne. Or c'est du matériel ancien qui roule sur la ligne entre

Lors de l'examen par notre assemblée, voilà quelques années, du projet de loi autorisant la ratification de l'accord franco-espagnol pour la réalisation de la ligne à grande vitesse transpyrénéenne Perpignan-Figueras, j'avais j'avais beaucoup insisté, en ma qualité de rapporteur, sur l'urgence qui s'attachait à réaliser concomitamment le tronçon Montpellier-Perpignan. Les années ont passé, la section internationale Perpignan-Figueras a bien été réalisée, mais

Plus récemment, et fort heureusement, les ministres des transports des précédents gouvernements avaient rassuré élus, populations et acteurs économiques quant à la volonté de l'État de réaliser cette ligne à grande vitesse.

entend-il réserver au projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse-Narbonne ? Je rappelle que le projet de LGV Montpellier-Perpignan représente non seulement un atout économique majeur pour l'essor et le développement de nos territoires, mais également un enjeu en matière de mobilité et de développement durable. La ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan et l'axe Bordeaux-Toulouse-Narbonne doivent offrir des liaisons structurantes entre les trois métropoles régionales que sont Montpellier, Barcelone et Toulouse. L'enjeu est non seulement local, régional et national, mais aussi aussi européen. La ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan constitue un véritable maillon stratégique sur le plus grand des axes de lignes à grande vitesse européennes. Le statut international de la ligne a été reconnu et il a été admis que son utilité et ses enjeux dépassaient largement ceux du seul tronçon considéré. Cette liaison rapide avec Barcelone et toute la Catalogne constitue un véritable levier économique pour l'eurorégion. La LGV Montpellier-Perpignan permettrait de garantir tant la continuité des réseaux à grande vitesse entre la France et l'Espagne que les énormes investissements déjà réalisés. Enfin, dois-je rappeler l'union sacrée des collectivités autour non seulement de ces deux projets de ligne à grande vitesse, mais aussi des modalités de desserte des agglomérations, dont la gare de Narbonne-Montredon. Allez-vous me rassurer, monsieur le secrétaire Allez-vous dissiper mes craintes ? Quelles sont les véritables intentions du Gouvernement sur ces deux dossiers majeurs ? La parole

Bordeaux-Toulouse-Narbonne, qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en 2016, représente quant à elle un investissement de 5,9 milliards d'euros. Ces deux projets nécessiteraient donc un investissement total d'au moins 10 milliards d'euros, qui devra être supporté exclusivement par la puissance publique. En effet, je le rappelle, la « règle d'or » empêche désormais SNCF Réseau de financer les nouveaux projets par sa dette,

a annoncé, le 1 juillet dernier, une pause de tous les grands projets d'infrastructures de transport. Mme la ministre chargée des transports, dont j'excuse à nouveau l'absence devant vous, a toujours eu une position claire sur le futur des mobilités : il faut reconstruire nos modes de pensée mais aussi nos solutions. C'est tout le sens de cette pause

Comment s'y prendre ? Il faut rechercher, d'abord, toutes les optimisations des réseaux existants qui peuvent redonner de la régularité et de la capacité à nos services de transports. C'est une nécessité que nos concitoyens attendent au quotidien. L'objectif,

pour les deux projets dont vous faites état, monsieur le sénateur, mais vous comprendrez que mon propos concerne l'ensemble des projets d'infrastructures que notre pays peut connaître. Quelle est la prochaine étape ? Les Assises de la mobilité et les travaux du Conseil d'orientation

depuis des décennies. Dois-je rappeler que la volonté de favoriser les échanges entre la France et l'Espagne s'est manifestée, en 1992, lors du sommet franco-espagnol d'Albi Elle a été réaffirmée lors du sommet de Tolède en 1993. Les deux gouvernements ont décidé la réalisation d'une ligne à grande vitesse à écartement international de Montpellier à Narbonne et Barcelone. Le sommet franco-espagnol de Foix, en 1994, a défini le tronçon de la liaison Paris-Madrid par Montpellier et Barcelone, qui irait de Barcelone à Narbonne, point d'où les futures lignes se dirigeraient vers Montpellier, Paris et Toulouse. Ce tronçon devait, en principe, être mis en service au cours de la période 2002-2005.

l'Europe du Nord au sud de l'Espagne, le seul maillon manquant. Voilà qui explique, monsieur le secrétaire d'État, notre exaspération.

quant à la réalisation pleine et entière du futur réseau Grand Paris Express, dont plusieurs lignes sont remises en cause, il fait preuve d'une obstination qui confine à l'absurde concernant le projet CDG Express. me faut d'abord faire remarquer que cette liaison privée aura pour l'usager un coût : le titre de transport est estimé aujourd'hui entre 27 et 29 euros et la tarification du STIF ne s'y appliquera pas. pas. Les infrastructures nécessaires à la réalisation de cette ligne privée reposent entièrement sur des deniers publics, car la société de projet est abondée en fonds propres par la SNCF et Aéroports de Paris. De source interne à SNCF Réseau, le coût global de ce projet est estimé aujourd'hui à 2,12 milliards d'euros. Pour autant, le CDG Express ne desservirait ni les arrondissements parisiens ni les villes de la banlieue parisienne qu'il traverserait.

En effet, le CDG Express utiliserait en grande partie le réseau ferré existant, alors que celui-ci est déjà saturé, ce qui ne manquera pas d'avoir des conséquences dramatiques pour les usagers des lignes B, E, H, K et P, pour ceux du TER Picardie et pour le fret. D'un point de vue environnemental- le secrétaire d'État à la transition écologique devrait être sensible à cet argument -, le CDG Express serait également néfaste. Cela est clair au vu des procédures d'expulsion d'extrême urgence qui concernent 29 hectares de terres agricoles de nouveaux tronçons au coeur d'une zone Natura 2000 ou encore de la dégradation de l'environnement urbain des habitants de la porte de la Chapelle à Paris, dont on connaît déjà l'état actuel et où le train passera 152 fois par jour sous les fenêtres des riverains.

Et l'impact financier sur les autres lignes reste à établir ! On le voit, le CDG Express est en exacte opposition à la priorité aux transports quotidiens affichée

comptes et d'autres -n'a manqué de souligner son impact négatif pour les transports du quotidien. Pas un seul n'a manqué de sommer le gestionnaire de fournir des garanties solides sur le sujet. À ce jour, aucune réponse nette et précise n'existe quant à ces questions primordiales. Monsieur le secrétaire d'État, en un mot comme en cent, ce projet reste inutile et coûteux. Il ne manquera pas d'avoir des conséquences désastreuses sur le transport quotidien des Franciliens. Il faut avoir le courage de l'abandonner. C'est l'engagement que j'attends de votre réponse.

je ne vais pas vous surprendre : le Gouvernement ne partage pas votre point de vue. Je doute de pouvoir vous convaincre, mais je vais tenter d'apaiser vos craintes. La qualité de cette liaison ferroviaire est vitale pour l'économie et pour l'attractivité de notre pays et de sa capitale, Paris, dont vous êtes sénateur et qui est la première destination touristique d'Europe. La nécessité de cette infrastructure nouvelle est donc établie

direct sur la pollution de l'air et le changement climatique en décongestionnant les voies rapides du nord de la région parisienne, qui en ont bien besoin. Par ailleurs, quant au confort des voyageurs, dans le RER, les voyageurs avec leurs bagages et les voyageurs du quotidien se gênent mutuellement. Il y a une forme de conflit d'usage, comme disent les techniciens des questions de transport. Cela est vrai,

en mars 2017 après un avis favorable de la commission d'enquête. Sa construction sera réalisée dans le cadre d'un montage juridique associant SNCF Réseau, Aéroports de Paris et la Caisse des dépôts et consignations. Je tiens, monsieur le sénateur, à vous préciser que le projet sera réalisé sans subventions publiques. Il ne pèsera donc pas sur les financements nécessaires à la modernisation du RER B, puisqu'il sera entièrement financé par la vente de billets sur cette liaison, donc par l'usager,

en faveur des transports du quotidien dans le cadre du nouveau contrat de plan 2015-2020. Une enveloppe totale de 7,5 milliards d'euros est prévue pour les projets de transports collectifs régionaux, dont près de 1,3 milliard d'euros pour les schémas directeurs des RER ; 230 millions d'euros ont d'ailleurs déjà été engagés, depuis 2015, Enfin, et toujours au profit des voyageurs du quotidien, il faut bien entendu mentionner la réalisation du Grand Paris Express, dont les travaux sont lancés au sud de Paris et qui viendra soulager les lignes existantes. Je doute de vous avoir convaincu, monsieur le sénateur, mais j'espère au moins vous avoir apaisé.

qui puisse me rassurer ou convaincre des acteurs attachés à la transition écologique. Ce projet est un non-sens de ce point de vue. Il causera des nuisances extraordinaires, il sera déséquilibré et l'investissement réalisé est démesuré et contraire à l'intérêt général. J'y insiste, reste une insulte- je pèse mes mots -à la dignité des habitants de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et du nord de Paris, qui verront cette ligne passer sous leurs yeux sans pouvoir y accéder. C'est même le cas des salariés très nombreux- plusieurs dizaines de milliers -de la plateforme aéroportuaire. Il est temps d'arrêter ce type d'aménagement qui ne bénéficie qu'à un très petit nombre d'usagers au détriment de l'immense majorité de ceux qui ont besoin d'une amélioration des transports. Il faut un autre projet : donner les moyens d'une forte accélération des investissements pour les lignes de RER et, plus particulièrement, pour la ligne B, qui dessert notamment l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Ces investissements pourraient être financés la création d'une recette dédiée, comme une augmentation de la taxe locale sur les bureaux, que nous proposons. Par ailleurs, l'une des solutions efficaces et à court terme qui permettrait de désengorger le réseau et, notamment, la ligne B serait d'augmenter la fréquence de la ligne K, ce qui requiert des moyens.

doubler le tunnel entre les stations Châtelet et Gare du Nord, ce qui permettrait d'absorber deux fois plus de trafic pour les RER B et D, et réaliser le bouclage du RER B entre Mitry-Claye et l'aéroport. Investir dans du matériel roulant neuf, comme cela a été fait sur d'autres lignes, ne serait sans doute pas de trop. Je vous encourage donc une nouvelle fois à suivre ces pistes plutôt que de vous entêter dans un projet contraire à l'intérêt général du point de vue tant financier qu'écologique.